Avec l'arrêt du 15 juillet dernier, c'est désormais l'ensemble des activités militaires qui se trouve menacé par la Cour de justice de l'Union européenne. Cet arrêt affirme que les militaires des États membres sont assujettis au même droit du travail que n'importe quel travailleur, exception faite des opérations. Cette décision introduit une notion de catégorisation. Il y aurait d'un côté des militaires qui combattent sur le terrain et ne sont pas soumis à la limitation du temps de travail et, de l'autre, tous ceux qui sont affectés à des fonctions de support ou à la préparation opérationnelle, dont le temps de travail va être encadré par le droit européen. Cet arrêt remet en cause le principe d'unicité du statut militaire en France et la doctrine selon laquelle les forces armées doivent être disponibles « en tout temps et en tout lieu Si l'on peut combattre sur le terrain, c'est parce que le matériel est bien entretenu et que l'approvisionnement est maîtrisé. C'est donc la sécurité même de nos militaires qui est en jeu, car pour être performant en opération il faut pouvoir se former et s'entraîner de manière bien spécifique. Madame la ministre, nous savons que vous avez conscience du problème posé par cet arrêt. L'application de cette décision annoncerait la fin de notre modèle d'armée complet et nécessiterait le recrutement de 30 000 militaires supplémentaires, ce qui est impensable

Enfin, pensez-vous que la Cour de justice de l'Union européenne puisse convaincre les groupes armés terroristes de passer, eux aussi, à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures entrecoupées de temps de repos compensateur ?

Tailler ainsi l'action militaire en morceaux n'est conforme ni à l'histoire de nos armées ni à l'ambition que nous portons pour elles. Le temps de travail des militaires ne se décompte pas, car c'est la réalisation de la mission qui prime. Depuis quatre ans, partout où je me suis rendue en France, je n'ai vu que des femmes et des hommes totalement engagés au service des Français. Depuis quatre ans, monsieur le sénateur, ni Florence Parly ni moi-même n'avons jamais été interpellées sur la question du temps de travail. Les militaires sont profondément attachés à leur statut, et le pays est profondément attaché à la disponibilité de nos forces armées. Nous sommes en train d'analyser précisément toutes les implications de cet arrêt de déterminer la meilleure réponse à lui apporter. S'il apparaît que la seule solution est de faire évoluer le droit applicable, c'est-à-dire la directive européenne sur le temps de travail, alors nous nous engagerons résolument dans cette voie, afin de permettre aux États membres qui le souhaitent d'exempter totalement leurs forces armées de son application. Il n'y aura pas en France une armée à deux vitesses ; c'est impossible. Je ne le souhaite pas, Florence Parly non plus, et je peux vous assurer que ni les militaires ni les Français ne le souhaitent.

Ce logiciel est développé par la société NSO, qui est contrôlée par le gouvernement israélien. Celui-ci propose les services de cette entreprise à d'autres États, de la même façon qu'il a vendu à l'Azerbaïdjan les drones de combat utilisés lors de son agression contre l'Arménie et la République d'Artsakh. Sur le théâtre des opérations de la guerre numérique, la société NSO agit comme un mercenaire du piratage. Elle achète sur un marché international des failles de sécurité qui peuvent se vendre plus d'un million de dollars et fournit ensuite à des gouvernements des programmes de surveillance. Des pays que l'on dit être nos alliés lui en ont acheté pour nous espionner : c'est le cas du Maroc. Ce marché du piratage, animé par des sociétés de mercenaires du numérique, ne pourrait exister sans l'activisme, la protection ou la passivité coupable des États. Monsieur le ministre, quelles actions la France va-t-elle entreprendre pour porter, sous l'autorité des organisations internationales, un projet de contrôle de ces activités ? Il existe une convention sur l'interdiction des mines antipersonnel ; de la même façon, nous avons besoin d'un traité international de non-prolifération de l'espionnage de masse pour protéger nos démocraties et nos libertés individuelles. La parole est

qui est opportune. J'ai aussi entendu vos propositions ; nous allons les examiner avec intérêt. Sur le fond, M. le Premier ministre s'est exprimé hier devant l'Assemblée nationale

M. Pierre Ouzoulias, pour la réplique. Pégase est né du sang de la gorgone Méduse, dont le regard pétrifiait les victimes. Face aux entreprises du numérique, votre gouvernement semble tout aussi paralysé Monsieur le ministre, agissez enfin pour défendre notre souveraineté numérique et notre indépendance nationale ! La parole est

mercredi dernier, la Commission européenne a présenté une série de mesures législatives destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne et à donner corps au Pacte vert européen. Si la route est encore longue avant que ces mesures ne deviennent réalité, elles sont spectaculaires et méritent indubitablement d'être saluées. Au même moment, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg, des pluies diluviennes ont provoqué l'une des pires catastrophes naturelles de ces cinquante dernières années. Le dernier bilan fait état de 165 morts en Allemagne et de 31 morts en Belgique. Les dégâts matériels sont considérables. S'il est encore trop tôt pour établir un lien direct entre le réchauffement climatique et ces inondations, nous savons en revanche qu'elles ont vocation à se multiplier et à s'intensifier dans les années à venir. La concomitance de ces deux événements nous rappelle cruellement, une fois encore, que la baisse des émissions de gaz à effet de serre ne saurait être notre seul horizon en matière climatique. Dans son rapport annuel, le Haut Conseil pour le climat recommande ainsi l'élaboration d'une stratégie nationale d'adaptation au réchauffement climatique ; il nous alerte ce faisant sur notre impréparation face à de tels risques.

Monsieur le ministre, quels enseignements tirez-vous de ces événements ? Disposons-nous de moyens suffisants pour les détecter- je pense notamment aux nouveaux supercalculateurs de Météo France -et pour prévenir les risques d'inondation ? quelle stratégie le Gouvernement envisage-t-il afin d'adapter nos territoires aux conséquences du réchauffement climatique et de nous éviter, autant que possible, de connaître dans l'Hexagone comme outre-mer une telle catastrophe ?

le sénateur Théophile, vous interrogez le Gouvernement sur les inondations survenues en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et dans le nord-est de la France. Permettez-moi avant tout d'exprimer au nom du Gouvernement notre soutien aux familles et aux États terriblement terriblement touchés par ces dramatiques événements, qui nous rappellent- vous l'avez dit -que le dérèglement climatique est déjà à l'oeuvre et que nous devons nous en protéger. Cela passe d'abord par davantage de prévention. Tel est l'objet des 200 plans que nous élaborons aux côtés des collectivités ; je pense notamment à ceux qui sont composés pour les 32 communes de la Guadeloupe, ou encore pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. Nous protéger impose également de développer nos capacités de prévision.

Monsieur le Premier ministre, dans cette pandémie qui n'en finit pas, le courage politique consisterait à dire à tous les Français qu'ils doivent obligatoirement se faire vacciner, quel que soit leur environnement professionnel. ce serait d'affirmer que se faire vacciner, c'est poser un acte de solidarité et même de fraternité, car c'est placer l'intérêt de l'autre au-delà de son intérêt propre et considérer l'individu, non pas comme une pièce unique et autocentrée, mais comme un citoyen conscient du rôle qu'il doit jouer dans un moment crucial pour le groupe auquel il appartient. ce serait d'assumer une décision de vaccination universelle obligatoire qui permettrait de ne pas fracturer la société française. En somme, ce serait l'exact inverse de ce que vous nous proposez Vous réduisez l'obligation à certaines professions ; elles sont certes très concernées par le virus, mais ne le sommes-nous pas tous ? Vous découpez l'espace public en lieux accessibles et non accessibles ; plus grave encore, vous demandez à des personnes privées de contrôler la situation sanitaire des individus. venez pourtant de découvrir, semble-t-il, que vous ne pourriez pas leur faire contrôler les identités sans remettre en cause les principes de liberté de circulation et d'anonymat constitutifs du pacte républicain. Vous voilà pris au piège : un contrôle de passe sanitaire sans contrôle d'identité ne vaut rien, mais un contrôle d'identité par des personnes non habilitées est impossible Une fois de plus, vous n'avez pas anticipé l'évolution du virus ; une fois de plus, cela vous conduit à prendre des mesures dans l'urgence, sans débat démocratique réel, des mesures qui entravent de plus en plus l'exercice des droits et des libertés des Français. Pensez-vous sincèrement que cela sera de nature à apaiser une société qui doit absolument l'être pour accepter le principe de la vaccination universelle ? Il est encore temps, mais allez-vous nous entendre ?

et des familles. Madame la sénatrice, loin des fractures de la société française que vous évoquez, laissez-moi vous dire que vous avez raison : la vaccination, ça marche ! D'ailleurs, les Français l'ont bien compris les Français l'ont bien compris : d'ici à la fin du mois de juillet, 40 millions de nos concitoyens auront bénéficié d'une première dose de vaccin. M. le Premier ministre l'avait annoncé pour la fin du mois d'août, mais c'est bien à la fin du mois de juillet que cet objectif sera atteint.

Ces derniers jours ont vu le contexte sanitaire se dégrader très rapidement, avec une hausse des contaminations de plus de 150 % par rapport à la semaine dernière. Cette situation entraîne la mise en place de nouvelles mesures, qui rendent dès aujourd'hui le vaccin plus que nécessaire pour la plupart de nos activités.

Monsieur le ministre, permettez-moi de rappeler que les semaines à venir vont être particulièrement difficiles dans nos établissements de santé et chez nos médecins généralistes en cette période de congés annuels. Chaque été, et plus encore cette année, les pénuries de personnel et la désertification médicale deviennent des maux du quotidien. On estime que 10 millions de Français vivent aujourd'hui sur un territoire où l'accès aux soins est difficile, sans qu'aucune mesure parvienne à stopper durablement l'hémorragie. La moitié des médecins de campagne ont plus de 55 ans. Cet été, dans un grand nombre de régions, faute de remplaçants en nombre suffisant, des cabinets médicaux devront fermer ; 50 % des offres de remplacement n'auraient pas encore trouvé preneur.

Après des années de manque de personnel et des mois de crise sanitaire et de plan blanc, les soignants sont épuisés et voient avec dépit leurs demandes de congés remises en cause. Ma question est donc la suivante que peut faire le Gouvernement, à court et moyen terme, pour renforcer l'attractivité des métiers du soin et assurer enfin un accès aux soins partout et pour tous, quelle que soit la période de l'année ? Où en est-on des mesures attendues pour lutter contre la désertification médicale ?

épidémique difficile que vous avez rappelé, les soignants vont effectivement être mobilisés une fois encore. Je veux rappeler que tous les gestes qu'accomplissent les citoyens

santé est pleinement mobilisé sur cette question : Olivier Véran a encore très récemment demandé aux agences régionales de santé de lui adresser des informations précises sur d'éventuelles fermetures et sur toutes difficultés, afin d'anticiper la situation. La parole est à M. Joël Labbé, pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

du dérèglement climatique et les catastrophes qu'il entraîne appellent des décisions politiques fortes et rapides. Pourtant, comme le Haut Conseil pour le climat et le Conseil d'État l'ont récemment rappelé, les mesures prises par la France sont loin d'être à la hauteur. Vous vous réjouissez de l'adoption du projet de loi Climat et résilience, mais ce texte ne permet en aucun cas

de réduire nos émissions de CO2 de 30 % d'ici à 2030, bien en dessous de nos objectifs. La déconnexion entre la gravité et l'urgence des enjeux, d'une part, et la teneur de nos débats

surtout dans les jeunes générations, qui prennent conscience de l'ampleur de l'urgence climatique à laquelle nous faisons face. Alors, monsieur le ministre, allez-vous enfin prendre des mesures fortes pour le climat ?

(SDIS) du département du Nord, mais aussi en mobilisant un hélicoptère Dragon et des sauveteurs aquatiques. Je veux d'ailleurs remercier ici l'ensemble des agents de secours mobilisés à cette occasion. Sur le fond des choses, j'ai déjà eu l'occasion de répondre à M. Théophile que nous agissons à la fois pour la protection et sur les causes des maux climatiques que vous avez pu citer, tout comme sur leurs conséquences. Concernant la protection, j'ai eu l'occasion d'évoquer les plans de prévention construits avec les collectivités,

Notre responsabilité est immense ; elle nous honore. Mais la protection du peuple français et la sécurité collective européenne ont un prix : l'engagement et la disponibilité en tout temps et en tout lieu des femmes et des hommes qui nous protègent au péril de leur vie. Par son arrêt du 15 juillet 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a étendu l'application de la directive européenne sur le temps de travail à certaines activités exercées par les militaires. Sont exclues les activités de formation et celles qui sont exécutées lors d'opérations militaires ou d'événements qualifiés d'exceptionnels. C'est un moindre mal ! Cette décision c'est le moins que l'on puisse dire ! -dans un contexte international où les tensions se multiplient et où de nombreux pays se réarment. Les conséquences d'une telle décision sont difficilement lisibles. Nous connaissons la position de Mme la ministre sur le sujet et saluons son énergie. Cependant, les impacts réels de cette décision sur notre modèle de défense ont-ils été identifiés ? Quelles sont les marges de manoeuvre de la France sur ce dossier, en particulier dans le cadre de la présidence du Conseil de l'Union qui débutera au mois de janvier prochain ?

Lagourgue, vous revenez sur une question qui a été posée précédemment et à laquelle ma collègue Geneviève Darrieussecq a apporté une réponse. Vous l'avez dit : cette directive européenne date de voilà presque vingt ans. Elle n'a fait l'objet d'aucune transposition et la France est loin d'être le seul pays en Europe à avoir adopté cette position. Notre modèle continue donc à s'appliquer depuis et, depuis vingt ans, nos forces armées conduisent des opérations extérieures, assurent quotidiennement la sécurité des Français sans que ce droit du travail pose de problème aux militaires en matière d'organisation de leur mission. Cette décision, qui vient fragmenter l'action militaire dans le temps, méconnaît

une puissance nucléaire et le seul pays de l'Union européenne membre du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle a donc une grande responsabilité dans le concert international et doit conserver toute l'agilité qu'implique cette place. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons avec la plus grande fermeté aux conséquences, évoquées dans cet hémicycle, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et je vous le dis sans ambages, monsieur le sénateur, puisque c'était l'objet de votre question : nous ferons le nécessaire sur le terrain du droit pour garantir que la France dispose librement de ses forces armées. La permanence de sa sécurité dans les airs, sur la mer, sous la mer, sur la terre et dans l'espace exige une organisation à laquelle

a annoncé un véritable succès de la diplomatie fiscale française, laquelle aurait obtenu de l'OCDE et du G20 la création d'un impôt sur les sociétés mondiales au taux de 15 %. Il avait d'ailleurs annoncé quelques semaines auparavant que ce taux serait de 21 % ; il annonce aujourd'hui que ce taux pourrait être supérieur à 15 % dans les années à venir. Pis encore, quelques jours après cette annonce, l'Union européenne révélait qu'elle allait elle-même renoncer à l'impôt sur le numérique, la fameuse taxe GAFA, sous la pression des États-Unis. Or le ministre Bruno Le Maire a annoncé, lui, que la France allait maintenir envers et contre tous cette taxe GAFA, nonobstant les pressions des États-Unis. Monsieur le ministre, compte tenu de cette grande confusion, sur un sujet aussi essentiel, nous avons besoin de connaître la vérité. C'est cette vérité que je demande aujourd'hui. La parole est à M. le ministre délégué chargé des comptes publics.

que le secteur du numérique devait être mis à juste contribution. C'est d'ailleurs ce qui a amené la France à prendre position et à proposer au Parlement, qui l'a accepté, le vote d'une taxe sur les géants du numérique. Nous avons toujours indiqué que cette taxe nationale serait maintenue en vigueur tant qu'il n'y aurait pas une taxe internationale ou, à défaut, communautaire. Nous avons fait en sorte, avec Bruno Le Maire et sous l'autorité du Premier ministre, dans toutes les discussions menées à l'échelon européen, de garder dans le panier de ressources propres de l'Union européenne non seulement les quotas carbone et les mécanismes d'ajustement aux frontières, mais aussi la perspective d'une taxe sur le numérique. La persévérance, c'est un combat de quatre ans pour faire en sorte que les règles de la fiscalité internationale soient modifiées tenant compte du fait que la seule présence physique dans un pays ne suffit pas à justifier la possibilité de taxer la valeur créée et pour faire en sorte d'adapter la fiscalité internationale au numérique. Nous avons remporté des combats, d'abord au G7, au sein de l'OCDE et, désormais, au G20. Ce sont ainsi 132 pays ou juridictions qui ont donné leur accord pour modifier leur droit et faire en sorte que cette taxation internationale soit possible. Elle s'appuie sur deux piliers : d'une part, la révision des règles de répartition du droit à lever l'impôt

Blanc, pour la réplique. Par votre réponse, monsieur le ministre, vous confirmez ce que nous ressentons tous, à savoir une communication excessive sur ce sujet. En communiquant sur cet impôt, vous cherchez à masquer l'absence de recettes réelles que vous pourriez faire sur des réformes de fond, notamment la réforme des retraites.

Républicains. En l'absence de Mme la ministre des armées, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Le 3 février dernier, j'étais à cette même place et j'alertais sur les risques que faisaient peser les conclusions de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne sur notre armée. La ministre des armées

Au mois d'avril dernier, avec Jean-Pierre Chevènement, j'ai publié une tribune dans la presse sur cette question : c'est « un coup mortel porté à notre défense », avertissions-nous. Nous implorions alors le Président de la République de défendre notre armée et de s'exprimer. La ministre des armées tout comme le chef de l'État n'ont eu de cesse de nous rassurer. Visiblement, le Gouvernement n'a aucune influence en Europe. Maintenant que la CJUE a tranché et témoigné de sa méconnaissance totale des spécificités de l'engagement militaire, il faut agir dans l'intérêt de notre pays et de l'Union européenne. Une possibilité s'offre au Président de la République : reprocher à la Cour d'avoir statué au-delà des compétences que lui attribuent les traités. C'était la solution que je suggérerais au mois de février dernier. Monsieur le Premier ministre, soutiendrez-vous cette proposition ?

de défense et vous connaissez aussi très bien l'Europe. Vous savez donc que la Cour de justice de l'Union européenne est indépendante et qu'il ne s'agit pas là de questions d'influence politique de la France en Europe. C'est une décision qui a été rendue par une juridiction indépendante. J'affirme de nouveau, dans ce débat, l'attachement de ce gouvernement à la construction européenne : nous voulons une Europe forte et efficace dans le respect de la compétence des États membres. Toutefois, je le dis sans détour : en matière d'organisation de ses forces armées, la France n'entend pas déléguer sa compétence. L'action militaire est collective, elle ne se résume pas à l'addition d'emplois du temps individuels. La fierté de nos militaires, c'est de faire primer la réalisation de la mission sur toute autre considération. La responsabilité des chefs militaires, c'est d'être attentifs à chaque instant à la santé et au moral de leurs soldats. Par conséquent, la responsabilité de l'État, c'est de garantir aux militaires les droits qu'ils méritent. Les militaires ont de lourdes obligations, qui font l'objet de compensations adaptées ; cela s'appelle le statut général des militaires, vous le connaissez bien. Cette organisation donne pleinement satisfaction, elle fait la fierté et l'admiration des Français. La Cour de justice de l'Union européenne a joué son rôle. Nous jouerons le nôtre une réponse au droit par le droit s'impose. Dès lors que les conséquences de cet arrêt auront été précisément analysées pour l'ensemble des forces armées, nous prendrons les initiatives qui s'imposent. Nous le ferons avec rigueur sans nous soustraire à nos responsabilités, qui sont, je le rappelle, d'assurer en tout temps et en tout lieu la sécurité des Français, de prendre acte des décisions de justice de l'Union européenne et, enfin, d'agir pour faire évoluer le droit de l'Union européenne si notre sécurité l'exige. Monsieur le secrétaire d'État, une fois de plus, sans vouloir vous contrarier, je note que vous évitez soigneusement de répondre à ma question. Il ne s'agit pas de savoir si la CJUE a joué son rôle. Elle ne l'a pas joué. La renégociation de la directive que vous évoquez dans toutes vos réponses est une option que j'ai soulevée au mois de février dernier. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est celle des juges de l'Union européenne, qui statuent au-delà de leur compétence et qui s'attaquent au paragraphe 2

le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il devient et le monde extrêmement dangereux dans lequel nous vivons. Il faut conclure, mon cher collègue ! Le Quai d'Orsay et l'Élysée ont soigneusement évité de faire pression sur l'Union européenne. Maintenant, nous vous demandons d'agir pour défendre les militaires : ils ont besoin de soutien, pas de mots.

nos passes sanitaires. Enfin, elle était lisible du point de vue des activités. Comment expliquer qu'il n'y ait pas besoin de passe sanitaire pour les lieux de culte, mais qu'il en faille un pour le cinéma, ou que, dans quelques semaines, les jeunes devront présenter un passe sanitaire pour aller au théâtre, mais pas pour aller au lycée

à lever le gage de l'article 40 pour que nous puissions discuter de nos amendements sur l'obligation vaccinale universelle ?

pour la réplique. Monsieur le secrétaire d'État, je ne vous ai pas demandé une dissertation sur le vaccin, la covid, les citoyens, les élus locaux ... J'ai posé une question claire : que pensez-vous faire pour que le Parlement puisse débattre des différentes options ? En particulier, êtes-vous prêt à lever le gage imposé par l'article 40

que l'obligation vaccinale est plus coûteuse pour l'État que votre système ? Si la réponse est oui, cela signifie que votre système ne vise pas à vacciner le maximum de Français. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour le groupe Les Républicains.

Sa réponse a été brève est limpide et c'est empreint de certitudes qu'il a assuré que plusieurs millions de doses étaient livrées chaque semaine. Vous avez ensuite précisé ses propos en annonçant l'existence d'un stock de 6 millions de doses, stocks auquel s'ajouteront, chaque semaine au mois d'août, 4,5 millions de doses. Nous disposerons donc, dans le mois à venir, de 24 millions de doses. Nul besoin d'être grand clerc, monsieur le Premier ministre : le compte n'y est pas pour atteindre votre objectif de 50 millions de vaccinés d'ici à la fin de l'été. Les doses manquent. Pour preuve, les mails de l'agence régionale de santé (ARS) à différents centres de vaccination dont je me contenterai de lire les grandes lignes, celles qui figurent en rouge et en lettres capitales : « Très très urgent. Problème d'approvisionnement en vaccins au niveau national. Nous sommes contraints de fermer la prise de rendez-vous pour des premières injections Doctolib et la plateforme téléphonique Monsieur le Premier ministre, loin de moi la volonté d'agiter les peurs, mais je m'interroge aujourd'hui, comme des millions de Français. Pourquoi annoncer le lundi 12 juillet l'application dans des délais très brefs du passe sanitaire avec un parcours vaccinal complet,

et nous attendons des approvisionnements de 2 millions de doses par semaine. L'objectif fixé par le Premier ministre que nous atteignions la primo-injection de 50 millions de nos concitoyens à la fin du mois d'août sera bien atteint, parce que nous disposerons

avec l'ensemble des professionnels de santé- je rappelle que le spectre les personnes pouvant vacciner a été élargi -, afin que nous puissions, durant l'été, procéder à l'ensemble de ces primo-injections pour nos concitoyens. La parole est à

La parole est à Mme Brigitte Devésa, pour le groupe Union Centriste.

M. Vincent Fichot, un Français originaire de mon département, les Bouches-du-Rhône, et vivant au Japon, est empêché de voir ses enfants depuis leur enlèvement par leur mère japonaise en 2018. Cela fait douze jours qu'il a entamé une grève de la faim dans la gare de Tokyo, à deux pas du stade olympique, et ce à quelques jours de l'arrivée d'Emmanuel Macron au Japon. La garde partagée des enfants en cas de séparation n'existe pas légalement au Japon. Aussi, l'enlèvement parental est une pratique courante et tolérée par les autorités locales. Il n'existe pas de chiffres officiels, mais des associations estiment que 150 000 mineurs en sont victimes chaque année dans l'archipel. Parmi eux, nombre de binationaux, dont les parents victimes, après s'être heurtés aux autorités et à la justice japonaises, se sont tournés vers les Nations unies. En 2019, ils ont porté plainte auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La justice française est également saisie. Une information judiciaire pour soustraction de mineurs visant l'épouse de notre compatriote en grève de la faim a été ouverte à la ans, M. Emmanuel Macron s'était engagé à agir en faveur de ces parents français, évoquant des « situations de détresse qui sont absolument inacceptables ». Au cours de sa visite au Japon, nous croyons savoir qu'il consultera le gouvernement japonais sur ce thème. pouvez-vous nous le confirmer et nous dire quelles actions diplomatiques sont prévues pour mettre fin à ces enlèvements parentaux ? La parole : quand les enfants sont au coeur d'un conflit familial, c'est toujours difficile, mais ça l'est particulièrement au Japon où, comme vous l'avez dit, le droit familial ne reconnaît pas l'autorité parentale partagée et où la non-présentation d'enfant ne constitue pas une infraction pénale.

d'exprimer nos inquiétudes sur cette situation. Régulièrement, nos services reçoivent des parents d'enfants franco-japonais qui font des demandes et nous intervenons régulièrement auprès des autorités japonaises, en particulier avec le président du collectif Sauvons nos enfants Japon.

sur ce dossier et nous sommes aujourd'hui en contact quotidien avec ce père de famille pour assurer un suivi de sa situation, notamment sur le plan médical, et lui apporter toute l'aide possible dans la limite de nos compétences. Naturellement, nous ne pouvons pas nous immiscer dans des procédures judiciaires qui concernent des conflits familiaux d'ordre privé, lorsque ces conflits ont lieu à l'intérieur même du Japon et qu'ils relèvent des seules juridictions locales, mais je peux vous assurer que cette situation fera partie des sujets qu'évoquera le Président de la République lors de son déplacement au Japon. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises, singulièrement dans cette configuration. Nous exprimons toute notre solidarité à M. Fichot et nous essaierons d'agir pour que

Vous avez eu raison de pointer les outrances et les images abjectes utilisées par certains extrémistes lors des manifestations contre l'obligation vaccinale et le passe sanitaire.

je vous pose donc la question : est-ce agir en responsabilité de fracturer l'unité du peuple français, qui est consacrée par notre Constitution, en dressant les vaccinés contre les non-vaccinés ? La

C'est raté ! Vous avez raison, certains entretiennent des fractures de façon artificielle ! Plus que jamais, mesdames, messieurs les sénateurs, notre pays a besoin d'unité.

des ministres. Heureusement ! C'est le rôle du Parlement que de l'améliorer, et j'espère, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous parviendrez à un texte satisfaisant, qui nous permettra, tous ensemble, de lutter efficacement contre la résurgence de l'épidémie.

Vous dites souvent que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Chers collègues, voulons-nous d'une société dans laquelle les droits sont différents selon les choix en conscience des citoyens ? Voulons-nous d'une société dans laquelle chacun pourra surveiller l'autre ? Je répondrai à ces questions par une citation d'un prix Nobel de la paix qui connaît bien le prix de la liberté, Nelson Mandela : « Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. » Nous sommes en train de nous attaquer aux fondements de notre société française, de notre trinité républicaine, « Liberté, Égalité, Fraternité », en sapant le premier, essentiel, la liberté. La

L'évolution actuelle et prévisible de la situation sanitaire dans les outre-mer inquiète légitimement. Partout, les taux d'incidence et de reproduction sont alarmants, et les capacités hospitalières restent sous-dimensionnées. Outre-mer, le taux de couverture vaccinale oscille entre 18 % et 32 %, soit trois fois moins que le taux national. La carte des plus faibles vaccinations recouvre parfaitement celle de la pauvreté, de l'accès aux services publics, des inégalités sociales et des fractures territoriales, éducationnelles et générationnelles. Derrière ces fractures, il y a une déficience de politique publique. La lutte contre la pandémie doit donc désormais se conjuguer à une lutte résolue contre ces inégalités. Si l'on ne peut reprocher au Gouvernement d'être demeuré inerte, il reste manifestement beaucoup à faire. Le passe sanitaire que vous nous imposez n'est pas, dans son économie, dans sa portée et dans son effectivité probable, de nature à endiguer l'épidémie et à nous rapprocher de l'objectif d'immunité collective, si ce n'est au prix de très graves atteintes aux libertés fondamentales et à la vie privée et professionnelle. Sur ces travées, nous pensons que seule la vaccination obligatoire, progressive, universelle et gratuite pour tous les adultes et le maintien de la gratuité des tests sont de nature à concilier les libertés individuelles et la sécurité sanitaire collective. Face aux réticences et aux oppositions, face à la peur et à la désinformation entretenues, quelles adaptations et quels moyens nouveaux comptez-vous engager pour véritablement aller vers les gens et, enfin, infléchir la mauvaise tendance outre-mer ?

... Le gage ! Il me semblait que la réponse du Premier ministre était assez claire à ce sujet ... Je pensais que vous alliez me parler de l'outre-mer et de la Guadeloupe, mais c'est peut-être ce que vous avez fait au début de votre question. Si vous me le permettez, je vais vous répondre sur cet aspect. La situation dans les outre-mer est effectivement

à vous faire vacciner sur l'île. Nous devons tout mettre en oeuvre afin que la population puisse se vacciner et se protéger contre la propagation extrêmement rapide du virus sur le territoire. La

gens. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour le groupe Les Républicains.

par des affrontements liés au trafic de stupéfiants : 600 clients par jour dans ce quartier, 80 000 euros par jour de chiffre d'affaires, et même 100 000 euros quand tout va bien ! La lutte contre ce trafic a enregistré de très bons résultats, puisque 30 kilos ont été saisis à Cavaillon, grâce au travail réalisé dans des conditions difficiles par les équipes de police,

La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour le groupe Les Républicains.

couacs sur la gratuité des tests, incertitudes sur le passe sanitaire ou le QR code ... Il aura fallu qu'avec mes collègues, Jacky Deromedi et Ronan Le Gleut notamment, nous intervenions encore et encore pour que les Français de l'étranger ne soient pas une énième fois traités comme des étrangers en France. Finalement, comme d'habitude, on bricole

Peine perdue : à ce jour, beaucoup de Français de l'étranger payent encore leur test en France. Les tweets, c'est bien, se faire obéir, c'est mieux ! Quant au passe sanitaire, vous avez annoncé le 13 juillet aux élus consulaires travailler à des solutions techniques afin d'obtenir un certificat pour tous les Français de l'étranger disposant d'un schéma vaccinal complet effectué avec un vaccin homologué ou un équivalent. Mais qu'entendez-vous par « un équivalent » Je vous ai écouté sur Public Sénat vendredi dernier. Le seul équivalent serait le Covishield. du Sinopharm, du Spoutnik et de bien d'autres ? de cette troisième dose que vous envisageriez L'été est déjà bien entamé, et beaucoup de nos compatriotes, début août, se verront appliquer des mesures encore plus contraignantes. Nous ne pouvons plus attendre, il faut des réponses concrètes et des solutions pour chacun. Alors, ma question est simple, vraiment simple : quand comment allez-vous faire des Français de l'étranger des Français à part entière, pour reprendre l'un de vos hashtags ? La parole est à M. le secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie.

examiner. Pour celles et ceux qui sont vaccinés avec des vaccins qui ne sont pas reconnus ou homologués par l'instance européenne, faute de données scientifiques probantes, suffisantes ou partagées,

la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Il va être

La séance est reprise. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public sur le projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

Une véritable déconcentration, susceptible de garantir une décentralisation, suppose inévitablement une présence renforcée, multipliée, des agents de l'État dans leurs différents métiers afin de soutenir

Deux crises fortes, l'une sociale- les « gilets jaunes » -et l'autre sanitaire, psychologique et économique, ont bouleversé et épuisé notre pays, mais elles ont aussi montré

car nous sentons que notre pays est un peu comme le temps : orageux et impétueux. Certains d'entre nous ont rêvé d'un grand soir de l'organisation territoriale, mais, les grands soirs étant parfois suivis de petits matins blêmes, nous avons pensé que ce n'était peut-être pas

à l'esprit français et cartésien de la norme, nous avons proposé un champ des possibles aux élus et des solutions selon un principe de subsidiarité : il faut que ce soit celui qui est le mieux placé

décousu, au cours duquel rien ne nous aura été épargné, tant sur la forme- réserves intempestives d'articles, mitage de l'examen jusqu'à une seconde délibération assez incongrue hier soir -que sur le fond. Le texte initial est le péché originel. Vous êtes pourtant connue, madame la ministre, pour être experte de notre système local et pour l'avoir fait progresser par de multiples initiatives. Quel contraste avec le texte que vous nous avez proposé !

Au-delà des correctifs mineurs, pour certains utiles, ce projet de loi comportait pour nous six écueils : une différenciation qui rate sa cible ; une décentralisation trop résiduelle une déconcentration ressemblant plus à une recentralisation ; une simplification complexificatrice- c'est un comble ! - ; un traitement lacunaire de la question des ressources financières des collectivités ; en dessert, l'ignorance totale de la question démocratique alors qu'elle aurait dû être une composante majeure.

compétences des régions en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle ; transfert à la carte des compétences facultatives au sein des EPCI ; renforcement du pouvoir réglementaire des régions dans l'attribution de certaines subventions et aides, Après avoir évité les nombreuses irrecevabilités, une quinzaine de nos amendements ont été adoptés : obligation pour le Premier ministre de répondre aux propositions d'adaptations législatives

rétablissement, auquel nous tenions, de l'expérimentation de la recentralisation du RSA ; expérimentation pour développer un système de transport sur d'anciennes voies ferrées. De grands pas en arrière

Alors que les EPCI incarnent un espace de coopération nécessaire pour les politiques publiques, ils sont systématiquement opposés aux communes, qui leur doivent pourtant une partie de leur salut. C'est probablement parce que nous avons un désaccord de fond sur le principe de solidarité que nous ne comprenons pas cette valorisation du repli sur soi. C'est également pour cette raison qu'à la délégation de compétences tous azimuts nous préférons la coopération interterritoriale. La majorité sénatoriale a ainsi fait le choix de revenir sur l'intérêt communautaire, par exemple en matière de zones d'activité, alors que ces dernières

La majorité sénatoriale est également toujours plus dure avec les faibles : prise en compte du patrimoine pour l'attribution du RSA, affectation de la PCH à d'autres charges, tentatives de modification de la loi SRU, même si elles ont été, il est vrai, contenues par la rapporteure par la rapporteure pour avis. Certaines expressions entendues dans cet hémicycle concernant le RSA- je pense au mot « rente » -gagneraient à disparaître des comptes rendus. En détournant les possibilités qu'offre le pouvoir réglementaire local, la droite sénatoriale a atteint deux objectifs : décrédibiliser le principe de différenciation et stigmatiser les plus précaires. Le pouvoir réglementaire doit permettre de faire mieux ou plus, pas de raboter des droits sociaux ou les politiques volontaristes en matière écologique. Dans le même ordre d'idée, l'article 50 rendait finalement possible l'échange de données pour lutter contre le non-recours aux droits sociaux, mesure que le groupe socialiste avait déjà proposée en juin

Sur ce sujet, quand l'exécutif est constamment dans la stratégie d'évitement, la majorité sénatoriale est, elle, aux abonnés absents. La démocratie représentative ne peut être exclusive de toute autre forme de participation. Le temps de la démocratie à éclipses a vécu.

Pour toutes ces raisons- refus de la solidarité territoriale, remise en cause de la question sociale et négation de la démocratie locale -, nous voterons contre ce texte. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour la réunion Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, dire que la montagne a accouché d'une souris La base choisie pour la décentralisation n'étant pas la commune, votre projet de loi n'entraîne aucun changement de structure, d'efficacité et de représentativité des Français. Vous n'avez fait que mélanger le jeu de cartes, mais le château de cartes reconstitué est toujours le même une citadelle imprenable, dans laquelle des élus sont barricadés et à laquelle les citoyens peuvent très difficilement accéder. À l'intérieur, on s'y perd comme dans un labyrinthe. Aucune amélioration n'est prévue en matière de consultation citoyenne, les choix territoriaux se font sans l'aval des intéressés : il manque à ce texte un quatrième D, pour démocratie. De plus, le contrat de mixité sociale fixant les objectifs à atteindre en matière de logements sociaux est signé entre le maire, le président de l'EPCI et le préfet. Le maire est donc minoritaire pour décider de la politique d'habitat et de logement sur son propre territoire de quoi accentuer le sentiment de dépossession des élus locaux et des habitants. Certains grands défenseurs des valeurs républicaines de la mixité sociale vont devoir passer de la théorie du vivre ensemble à la réalité du « vivre avec Je leur souhaite beaucoup de courage et d'abnégation républicaine ! Les maires ne semblent pas vraiment être au centre de l'attention du Parlement, puisque la commission mixte paritaire sur le projet de loi Climat et résilience leur a refusé un droit de veto sur tout projet éolien envisagé dans leur commune. J'espère que l'ajout de cette disposition dans le présent projet de loi sera, lui, conservé à terme. Concernant plus particulièrement la métropole Aix-Marseille-Provence, les sénateurs de la majorité de droite ont défendu leur baronnie métropolitaine en laissant- bons seigneurs ! quatre-vingt-douze communes qui la composent, mais en rappelant bien que les compétences déléguées devaient rester sous la coupe souveraine de sa présidente, Martine Vassal.

à l'ogre métropolitain ! Qu'elles soient assurées de mon soutien dans leur résistance à l'oppression et à l'intégration de force. Oui, les citoyens et les élus locaux ont été chamboulés par les lois RCT, NOTRe et Maptam, mais il faudra à l'avenir remettre courageusement les choses à l'endroit en s'appuyant sur le triptyque commune-département-État. C'est là la clé d'une réelle « différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification ». La liberté et la subsidiarité sont nécessaires au respect des identités et à l'efficacité de l'action publique. Pour nos maires, premiers représentants et premiers acteurs de l'État décentralisé, il ne restera qu'un D, celui, pour rester poli, de débrouille. Des communes les plus rurales aux communes urbaines, petites et moyennes, chaque crise est gérée selon le système D, et ce texte n'y changera rien. Pour conclure, j'indique en faveur de ce petit texte pour appuyer les quelques possibilités introduites sur le renforcement du contrôle du versement du RSA, sur les délégations de compétences des métropoles aux communes, sur la libre autonomie municipale en matière d'éolien, en espérant, car je reste un éternel optimiste, que l'Assemblée nationale ne jouera pas les godillots du Gouvernement en cassant ces apports souhaités par les élus locaux. La parole est à M. Stéphane Le Rudulier, pour le groupe Les Républicains. Madame la

l'importance et la primauté de ces sujets, malgré les impératifs calendaires. Je m'adresse donc à vous avec beaucoup de respect, et je me réjouis de votre force de conviction, compte tenu du cadre contraint qui vous a été fixé par le Premier ministre et le Président de la République. Néanmoins, force est de constater que le texte initial n'était pas du tout à la hauteur de nos attentes, alors même qu'il nous avait été présenté comme le troisième acte majeur de la décentralisation.

lequel ne cesse de prospérer à travers notamment la multiplication des normes, l'organisation de la dépendance financière des collectivités et l'éloignement des principaux centres de décision des territoires ? Alors, oui, ce texte fut une réelle déception pour notre famille politique, car il manquait d'ambition à bien des égards, car il privilégiait généralement les mesures paramétriques, sous prétexte de simplification, tout en évitant de s'aventurer sur d'autres terrains essentiels, car il abordait de multiples sujets trop variés, qui auraient mérité à eux seuls un projet de loi. De De surcroît, ce qui a d'autant plus limité la portée du texte est bien évidemment l'absence d'un volet financier robuste, indispensable à une véritable décentralisation et à une différenciation. Pour autant, le Sénat ne s'est pas résigné. C'est avec une ferme intention de redonner corps à ce projet de loi que la Haute Assemblée a commencé ses travaux. Je voudrais saluer nos rapporteurs, qui se sont efforcés d'insuffler un surcroît d'ambition et d'envergure au texte. Je pense principalement

nous nous sommes appuyés sur les réflexions antérieures de la Haute Chambre. Je pense notamment aux fameuses 50 propositions du Sénat, qui ont été formulées sous la direction du président Larcher et remises au mois

Ainsi, le texte des commissions présentait déjà un certain nombre d'avancées. Je ne vais pas faire l'inventaire exhaustif de l'ensemble des apports du Sénat. Je souhaite néanmoins m'arrêter sur quelques mesures phares, notamment celles visant à garantir la possibilité d'un exercice différencié des compétences au sein du bloc communal par le biais du transfert « à la carte » de compétences, compétences, la suppression du caractère obligatoire du transfert des compétences « eau » et « assainissement » et de la gestion des eaux pluviales urbaines ou encore la consécration du principe selon lequel toute décision prise à l'échelon territorial relève prioritairement du préfet de département. Ces dispositions viennent parfaire le volet différenciation et déconcentration du projet de loi. Sur le sujet ô combien sensible du logement, le Sénat a adopté des mesures visant à permettre une meilleure conciliation entre l'action des collectivités et la réalisation des objectifs de la loi dite SRU, avec la prolongation du dispositif sans date butoir et en rattrapage glissant, la mise en place d'un rattrapage différencié et contractualisé un contrat de mixité sociale dont le maire et le préfet seraient la cheville ouvrière, ouvrant ainsi une démarche partenariale permettant de sortir du climat de défiance qui s'était installé depuis plusieurs années entre l'État et les communes carencées ou déficitaires, ou encore la suppression de sanctions inefficaces et contre-productives pour initier un système de fléchage des éventuelles pénalités de carence vers de la construction de logements. Sur le volet sanitaire et social, j'évoquerai la réforme de la gouvernance des ARS, qui se veut plus équilibrée à l'égard des élus locaux, laissant notamment la place à une coprésidence du préfet de région et du président du conseil régional.

depuis cinq ans du fait principalement d'une mauvaise répartition des compétences entre les différents échelons. J'insiste sur un point : le fait de revenir à l'esprit originel de l'intercommunalité constitue, je le pense, un véritable tournant historique, qui va permettre de rendre la parole aux élus locaux, afin de définir ce nouveau cadre institutionnel. Je voudrais saluer une nouvelle fois la qualité du dialogue que nous avons eu avec Mme la ministre sur ce sujet aussi essentiel pour le quotidien de 1,8 million d'habitants. Enfin, outre tous ces apports en commission, de très nombreuses dispositions comportant différentes améliorations et des éléments de précision du texte des commissions ont été adoptées en séance durant ces derniers jours. Nous espérons dès lors que l'Assemblée nationale saura se saisir de cette loi 3DS revigorée et nous accompagner dans une démarche de décentralisation qui se veut ambitieuse, en vue d'aboutir à une réelle consolidation des libertés locales.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, Chaque révolution s'évapore en laissant seulement derrière elle le dépôt d'une nouvelle bureaucratie », écrivait Kafka. Depuis plusieurs semaines, vous expliquez, madame la ministre, que ce texte n'est pas une révolution. C'est effectivement ce que nous constatons. Je ne sais si vous prendrez ce jugement comme un éloge ou comme une critique. Il y a, pour tout dire, un peu des deux. En tout cas, on peut approuver le fait que vous ayez évité à nos élus locaux et à nos concitoyens un nouveau bouleversement ; il n'aurait pas manqué d'apporter avec lui son lot de complexités administratives, dont les collectivités territoriales souffrent déjà trop. Je tiens à souligner la qualité de nos débats et à saluer nos collègues rapporteurs. Malgré un contexte délicat et un temps d'examen réduit, notre chambre a substantiellement enrichi le texte. Nous avons ainsi eu l'occasion de voter plusieurs dispositions visant à accroître la liberté des collectivités territoriales. Le rétablissement de l'expérimentation de la recentralisation du RSA, proposé notamment par notre groupe, a été adopté par le Sénat. Pour de nombreux départements, et pas seulement celui de la Seine-Saint-Denis, le RSA est une charge majeure qui pèse considérablement sur les budgets. Nous saluons également le renforcement du rôle du département en matière d'aide sociale et du poids des élus locaux au sein des conseils d'administration des ARS, ce qui permettra aux collectivités d'avoir une meilleure maîtrise de ces politiques. Nous soutenons à cet égard des élargissements du pouvoir réglementaire local portés par le texte, même s'ils sont modestes. Le texte comporte aussi un volet important sur le logement, qui aurait d'ailleurs pu faire l'objet d'un véhicule législatif à part entière. C'est l'un des sujets les plus importants pour les élus locaux, confrontés en permanence aux complexités de la loi SRU, à ses obligations, à ses seuils et à ses dérogations. Les contrats de mixité sociale apporteront des solutions adaptées aux réalités locales. Les communes qui ne respectent pas les obligations en matière de logements sociaux ne sont pas toujours des ennemis de la mixité sociale. Même si certains maires le sont, la plupart font de leur mieux pour composer avec les règles très rigides de la loi SRU. Ce projet de loi tel qu'amendé par le Sénat apportera davantage de souplesse et de liberté aux maires pour adapter le parc de logements aux objectifs fixés à l'échelle nationale. Partageant cette volonté de donner plus de souplesse et de liberté aux acteurs du terrain, notre collègue Emmanuel Capus a déposé un amendement tendant à modifier la loi SRU en rendant plus progressive l'entrée dans le régime d'obligation concernant les seuils de logements sociaux. Notre chambre a compris tout l'intérêt de ce dispositif pour les communes, et elle l'a adopté. Le texte apporte aussi de la souplesse aux opérations de revitalisation des territoires. Je veux notamment mentionner l'accélération de la procédure d'acquisition de biens sans maître, qui était attendue par les maires de petites communes Au fil de l'examen, les prérogatives des organismes fonciers solidaires ont été renforcées par le texte. C'est un point important pour l'aménagement de nos territoires. Grâce à l'adoption d'un amendement déposé par notre collègue Daniel Chasseing, les communes touristiques membres d'une communauté d'agglomération qui le souhaiteraient pourront désormais retrouver l'exercice de la compétence de promotion du tourisme. Pour faciliter la transition écologique dans nos territoires, il était nécessaire de clarifier les compétences des régions et des départements en la matière. Le maire se voit quant à lui confier la possibilité de réglementer l'accès aux espaces naturels protégés qui seraient menacés par une hyperfréquentation, ainsi que le souhaitait notre ancien collègue Jérôme Bignon.

Il est cependant arrivé qu'il s'entrave lui-même. Nous regrettons ainsi qu'un grand nombre d'amendements n'aient pas pu être examinés en raison d'une interprétation extensive de l'article 40 de la Constitution. Au motif que les transferts de compétences entre collectivités territoriales créeraient ou aggraveraient une charge publique, ils ont été déclarés irrecevables. Il y a plus de trente-cinq ans, le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui laisse effectivement penser que l'article 40 s'y opposerait. L'idée que la représentation nationale ne pourrait pas proposer par voie d'amendement un transfert de compétences entre collectivités territoriales est pour le moins étonnante. Or les parlementaires tiennent à leur liberté d'amendement. Par ailleurs, durant les trente-cinq ans qui nous séparent de la décision du Conseil Constitutionnel, la démonstration de la bonne gestion des deniers publics par les collectivités locales a été amplement apportée. L'État, quant à lui, a démontré l'inverse sur la même période et se garde bien de s'appliquer une règle similaire à celle de l'article 40. Nous sommes également nombreux à regretter l'application à géométrie variable de l'autre faucheur d'amendements : l'article 45 de la Constitution. Alors que le projet de loi 3DS entend simplifier l'action publique locale, les amendements de notre collègue Dany Wattebled, qui visaient à donner son plein effet au principe selon lequel « silence vaut acceptation », ont été déclarés, eux aussi, irrecevables. Ce mécanisme, selon lequel silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation, est essentiel pour nos concitoyens, nos élus et nos entrepreneurs. Il est aujourd'hui vidé de sa substance par une liste infinie de dérogations. Alors que nous avions l'occasion de remédier à cela en votant des dispositions déjà adoptées par le Sénat lors de l'examen du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, ces amendements ont été déclarés irrecevables sans aucune explication. Nous le regrettons vivement. Le texte comporte néanmoins plusieurs mesures de simplification qu'il convient de saluer, notamment celle qui prévoit le renforcement des échanges de données entre administrations, ainsi qu'entre Nos élus ont besoin de plus de simplicité, mais aussi de plus de soutien. Le projet de loi y répond en faisant du Cerema un outil au service de l'ingénierie territoriale de l'État et des collectivités. Ces dernières seront désormais représentées au sein de sa gouvernance. Dans ce même esprit, les chambres régionales des comptes verront leurs missions évoluer, afin d'ajouter à leur fonction de contrôle une assistance aux collectivités territoriales dans l'évaluation des politiques publiques. Au total, même si, comme je l'ai expliqué, nous regrettons que certains de nos amendements, que nous considérions importants, n'aient pas été pris en compte et même si les changements apportés par ce texte restent mesurés, nous pensons que celui-ci apporte des améliorations intéressantes à l'activité des collectivités territoriales. Le groupe Les Indépendants votera donc majoritairement en faveur de son adoption. La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

dire que la montagne a accouché d'une souris ne serait pas le plus approprié au vu de l'évolution du texte après son examen au sein de notre assemblée ; ou alors, ce serait une grosse souris ! En effet, En effet, si le texte initial était pauvre, souvent imprécis, quelquefois incohérent, nous voici à l'arrivée avec près du double d'articles, et ce malgré une grande libéralité, très souvent dénoncée dans l'hémicycle, dans l'application de l'article 40

Que dire donc ? Si les promesses de grand soir formulées lors du tour de France présidentiel après la crise des « gilets jaunes » ne sont pas au rendez-vous, après être partis d'un projet de loi n'apportant que des réponses parcellaires aux enjeux si importants de l'organisation territoriale de notre pays, nous arrivons à un texte qui ne brille pas par la cohérence des positions retenues. Nos positions, à nous, écologistes, sont stables depuis des années : « du local au global La crise des « gilets jaunes » et la crise sanitaire, dont nous ne sommes toujours pas sortis, ont rappelé l'attachement des Français et du pays à un échelon local plus souple, plus agile pour répondre à leurs attentes. Face à de nouveaux records d'abstention électorale, nous aurions pu saisir l'occasion pour innover et faciliter l'engagement des citoyens. Encore eût-il fallu en avoir le temps Pourtant, le texte tel qu'il résulte de nos débats ne consacre aucune nouvelle décentralisation, pas plus qu'une mise en oeuvre d'une différenciation efficace, sans parler d'une quelconque simplification On décentralise en reconcentrant ou on recentralise en déconcentrant. Et sans pouvoir répondre à la question des citoyens : « Comment ça marche ?

Aucune des propositions de notre groupe renforçant la démocratie locale ou le droit de pétition n'a été retenue, pas plus que le renforcement réel du pouvoir réglementaire du maire pour protéger la santé de ses administrés, ainsi que l'environnement. Pourquoi avoir autant peur, chers collègues, de la démocratie participative, qui ne nie pas l'élu et le pouvoir de ce dernier, mais vient le renforcer ? Limiter le droit de pétition et rendre optionnelle son inscription à l'ordre du jour d'un conseil municipal, c'est véritablement planter un couteau dans le dos du pacte républicain.

d'hypocrisie du positionnement majoritaire, qui consiste à donner un pouvoir de veto au maire pour l'implantation des éoliennes, structurant la politique énergétique de toute une région, tout en lui refusant le droit de réglementer les épandages de produits phytosanitaires pour protéger les habitants et les terres de son village.

Que dire aussi des possibilités offertes par la nouvelle rédaction de modifier sous couvert de simplification la portée des réglementations, notamment en matière d'aide sociale ou d'urbanisme ? J'ai eu l'occasion d'argumenter sur ce point : la simplification ne doit pas être synonyme de moins-disance. Essayons de rester positifs. Je salue le réveil de notre assemblée suite aux débats en commission sur plusieurs points : la suppression des mesures faisant du Ceser une chambre soumise à des nominations politiques, voire politiciennes locales, la possibilité d'expérimentation de la recentralisation du RSA ou une plus grande démocratie sanitaire, avec la participation accrue des citoyens, mais aussi des élus. Le titre relatif à la transition écologique, à l'instar de la loi Climat ou de la modification de l'article 1 de la Constitution, d'ailleurs non aboutie, n'est pas à la hauteur des enjeux. Quant à la remise sous coupe préfectorale de l'Ademe, une agence qui a fait ses preuves dans le domaine de l'environnement, elle laisse encore perplexes les intéressés et tous ceux qui ont bénéficié du soutien de cette dernière. Une fois passée la surprise de voir réapparaître un volet logement initialement prévu pour la loi dite « séparatisme », nous avons constaté que ni le Gouvernement ni cette majorité n'avaient à coeur de combattre l'assignation à résidence des populations précaires qu'ils dénoncent pourtant tant de fois. Tout comme pour les éoliennes, la théorie du « Pas chez moi » revient de plus belle. Comment justifier auprès de nos concitoyens la possibilité pour les communes de comptabiliser des casernes militaires comme logements sociaux ? Autres exemples de cette lutte contre les précaires plus que contre la précarité : le renforcement du contrôle des allocataires du RSA ou le refus de pérenniser l'encadrement des loyers.

voire avec une ambition trop partisane. Il ne permet notamment pas à la ville de Marseille d'être maîtresse de ses politiques de proximité, comme le sont les autres communes des Bouches-du-Rhône. Cette disposition devra donc être retravaillée rapidement et sérieusement. et sérieusement. Chers collègues, si je regrettais la timidité du Gouvernement, qui n'aura pas saisi l'occasion et qui a tardé à faire de réelles propositions pour un nouveau pacte territorial, je déplore aussi que la majorité sénatoriale ait choisi de se contenter de reprendre la vision partielle et quelquefois partiale de ses propositions antérieures sans aucune ouverture. Ce texte très étoffé, sans vision réelle structurante, sans cohérence dans le rôle de chaque échelon, ne résoudra pas les problèmes d'organisation et de coordination des communes, des métropoles et des régions. C'est pourquoi, quoique fervent défenseur d'une décentralisation à la hauteur des spécificités locales et d'une différenciation synonyme d'efficacité et non de compétition et d'inégalités,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, après trois semaines de travail et de débats nourris, la chambre des territoires a achevé hier soir l'examen du projet de loi dit 3DS. Fruit d'une longue gestation et de plusieurs mois de concertation, le texte porté par Mme la ministre Jacqueline Gourault, que nous saluons de nouveau pour l'immense travail réalisé, vient compléter les actes de décentralisation, qui- n'hésitons pas à le dire -ont parfois laissé des imperfections et des carences dans l'organisation actuelle de notre millefeuille territorial. En plus de répondre aux attentes pragmatiques qui ont été exprimées à plusieurs occasions, le projet de loi 3DS marque un tournant dans les relations entre l'État et les collectivités. Le texte s'appuie notamment sur la contractualisation, avec des outils concrets pour permettre aux élus locaux et aux collectivités territoriales d'exercer les missions qui sont les leurs, avec plus de risques, de responsabilités et de singularités. Ce texte se doit de tirer les leçons de la crise sanitaire en confortant le rôle des élus locaux et en améliorant la collaboration avec les services déconcentrés de l'État. Pour répondre à ces objectifs, le Gouvernement a proposé au Sénat un texte initial de reposant sur un juste équilibre entre les attentes légitimes des territoires et des élus locaux, largement consultés tout au long de la fabrication du projet de loi, sans bouleversement des équilibres existants. Après de nombreuses heures de débats, il faut noter le maintien des quatre-vingt-quatre articles de départ avec quelques modifications du Sénat, comme la décentralisation des routes aux départements, aux métropoles et aux régions qui le souhaitent, la mise en oeuvre différenciée et adaptée aux réalités locales des objectifs de la loi SRU, réforme qui n'avait jamais été envisagée durant les quinquennats précédents depuis le vote de la loi en 2000, le financement des établissements de santé par les collectivités et leur capacité de recruter des soignants pour leurs centres de santé, et même l'expérimentation de la recentralisation du RSA par l'État. Cela témoigne bien de l'écoute, de la compréhension et de la traduction législative des attentes concrètes de nos élus dans le texte du Gouvernement, modifié par le Sénat. Aussi, dans une ambiance constructive et sereine, grâce à l'esprit de compromis de nos rapporteurs, que je salue pour la qualité du travail réalisé, et pour le plein exercice des libertés locales, les sénateurs ont enrichi le texte, qui compte aujourd'hui plus de 200 articles.

groupes. Sur le titre relatif à la différenciation territoriale, nous nous sommes entendus sur l'extension du pouvoir réglementaire local, afin de développer les libertés locales, sur la suppression de la définition de la composition du Ceser par délibération du conseil régional le renforcement de la participation citoyenne locale, qui était très attendu par nos concitoyens. Concernant le titre sur la transition écologique, après de nombreux débats, nous sommes tombés d'accord sur le transfert des routes aux départements, métropoles et, à titre expérimental, aux régions volontaires- cas de la région Grand Est -, avec une version de compromis trouvée entre les rapporteurs et le Gouvernement, sur le transfert des petites lignes ferroviaires de manière plus encadrée ou encore sur les sanctions sur le domaine public fluvial géré par Voies navigables de France. le volet relatif au logement et à l'urbanisme, notre groupe a été particulièrement actif, afin de bien rappeler les difficultés auxquelles se heurtent nos élus locaux, notamment sur les atteintes des objectifs de la loi SRU. Vous avez d'ailleurs bien voulu adopter nos propositions sur l'augmentation des catégories de dépenses déductibles du prélèvement SRU et sur la possibilité accordée aux communes nouvelles de demander la conclusion d'un contrat de mixité sociale. En dépit de quelques divergences d'opinions sur des dispositions techniques, sur lesquelles nous resterons très attentifs dans le cadre de la navette parlementaire, sans dogmatisme, mais avec réalisme, nous nous sommes entendus sur la suppression de la date butoir de 2025 ou encore sur le rythme de rattrapage du déficit de logements sociaux différencié selon les communes SRU. Le Le titre relatif à la santé aura également nourri nos nombreux débats. Nous avons toutefois convergé sur une meilleure représentation des élus locaux au sein du conseil d'administration des ARS ou sur la participation des usagers dans les conseils territoriaux de santé et dans les contrats locaux de santé. Toujours sur ce titre, vous avez bien voulu adopter notre amendement facilitant l'implantation d'officines de pharmacies à Mayotte, afin d'assurer un meilleur maillage territorial en matière de santé. Les échanges sur Les échanges sur le titre relatif à l'outre-mer ont également été fructueux. Ils ont permis à notre groupe de proposer à la Haute Assemblée plusieurs dispositions attendues par les territoires ultramarins. Nous pouvons évoquer la mise à jour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les les conditions de la prescription acquisitive immobilière à Mayotte, la dérogation au code de l'urbanisme pour la construction de logements en Guyane, le statut de Clipperton ... C'est important ! ... ou encore la composition du congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe. La meilleure mise en oeuvre du service public numérique pour tous les usagers, avec l'application « dites-le-nous une fois », principe qui prévoit que les usagers n'aient plus à communiquer de nouveau les documents et informations que l'administration leur a déjà demandés par ailleurs, la faculté des collectivités et de leurs groupements de recourir au financement participatif pour leurs investissements ou encore l'extension du dispositif de réunion par visioconférence pour les conseils départementaux régionaux aux conseils des syndicats intercommunaux et aux syndicats mixtes fermés font partie des mesures de simplification qui ont été adoptées au Sénat. En conséquence, chers collègues, vous l'aurez compris, en prenant en compte ces éléments, le groupe RDPI votera en faveur du projet de loi 3DS, dans le droit fil des actions menées depuis 2017 en faveur des élus locaux et des collectivités. Nous émettons toutefois plusieurs réserves sur certaines dispositions adoptées par le Sénat. Si certains ont souhaité rejouer le match de la loi Engagement et proximité ou du projet de loi Climat et résilience, nous ne pouvons pas revenir sur les équilibres qui ont pu être trouvés, comme nous l'avions indiqué au début de l'examen.

ou encore l'obligation d'un avis conforme du conseil municipal pour les projets d'installation d'éoliennes sont des propositions que nous pouvons entendre, mais qui ne créent à ce jour aucun consensus et que notre groupe ne partage pas.

nous achevons quinze jours d'examen d'un projet de loi dont les débats furent finalement plus engagés qu'attendu, même s'ils furent toutefois sous-tendus par la fatigue du marathon législatif particulièrement intense que nous avons subi cette année. À cela s'ajoute l'amer constat, quasi unanimement souligné lors de la discussion générale, de voir combien ce texte, en arrivant sur nos pupitres, nous a paru éloigné de son ambition initiale et des fortes attentes qu'il suscitait de la part des collectivités, d'autant que son examen a suivi de quelques jours un scrutin marqué par une abstention record et préoccupante. Face à cet horizon encombré, le Sénat a toutefois su faire remonter toute la profondeur des problématiques locales. Nos échanges ont traduit combien la vie de nos territoires était riche que s'y jouaient des questions majeures de la vie de notre nation. Je pense, par exemple, à nos discussions autour de l'article 17 et de l'application de la loi SRU. Certains ont fait part de leur crainte que ce projet de loi ne dénature l'esprit initial de la loi au motif de davantage de souplesse. D'autres ont pu souligner, au contraire, qu'à défaut de souplesse, les objectifs de la loi SRU ne seraient jamais atteints, car parfois irréalisables. Néanmoins, au-delà des positions soutenues, nous nous accordons à regretter qu'un tel sujet n'ait pas fait l'objet d'une discussion à part entière, au lieu de le traiter entre le transfert des compétences « voiries » et la réforme de la gouvernance des ARS. Au cours des débats, certaines mesures adoptées ont révélé des clivages profonds mettant en lumière, là aussi, toute l'importance de la vie politique locale. le cas, par exemple, de la disposition adoptée en commission des lois qui permet au département de décider de priver du RSA les personnes disposant d'une épargne trop importante. Une majorité des membres du RDSE doutent que cette mesure soit la plus à même de lutter efficacement contre les abus de notre système de solidarité. solidarité. Nonobstant ces premières considérations, je veux saluer le travail du Sénat, à commencer par celui de nos rapporteurs. Notre assemblée a su non seulement s'approprier pleinement un texte au sujet duquel nous avions d'abord fait part de notre déception, mais aussi garder sa cohérence. C'est le cas de la réintroduction d'un droit à l'erreur pour les collectivités locales, qui, hélas ! peine toujours à vous convaincre, madame la ministre. Le groupe du RDSE tient également à saluer la transposition, dans ce texte, de la proposition de loi visant à moderniser et faciliter la procédure d'expropriation de biens en état d'abandon manifeste, largement adoptée au Sénat le 14 avril dernier, avec un avis favorable du Gouvernement. Ces dispositions devraient permettre de mieux soutenir la revitalisation de nos communes face au problème croissant de la sous-optimisation des biens immobiliers et des terrains abandonnés par leurs propriétaires. Malgré tout, je crains que nous n'ayons pas pleinement su rattraper les défauts et les insuffisances initialement constatés dans le volet de la différenciation, et cela malgré les améliorations apportées au cours de cet examen. de cet examen. La question de la portée réelle de ce principe se pose toujours, notamment au regard des moyens, d'autant que la différenciation porte en elle-même le risque d'une inégalité territoriale qui se creuserait encore davantage avec le temps. Si nous voulons que ce nouveau souffle territorial soit porteur d'un meilleur avenir pour nos collectivités, il faudra se montrer particulièrement vigilant dans les années à venir pour éviter toute forme de dérives et de particularismes locaux au détriment des territoires moins favorisés.

permettre aux communes touristiques membres d'une communauté d'agglomération de retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme ». Nos débats nous auront aussi permis d'éviter de commettre certaines erreurs, comme sur la modification de la composition des Ceser, à travers un amendement que je portais au nom de mon groupe. J'aimerais revenir sur la non-suppression de l'article 7 du projet de loi, qui institue une expérimentation permettant aux régions d'exercer la compétence d'aménagement et de gestion des routes nationales et autoroutes non concédées. Nous avons dit combien cette disposition nous interrogeait quant à la lisibilité des compétences des collectivités en matière de voirie routière, d'autant que les départements sont connus et reconnus pour l'exploitation de leur domaine routier, alors que les régions sont loin de disposer de telles compétences. Aussi, je regrette que cet article n'ait finalement pas été supprimé à la faveur d'un second vote, à minuit et demi, hier soir, alors que l'amendement que je portais avait été adopté dans la semaine. Pour l'essentiel, notre groupe demeure attaché aux communes et aux départements et ne souhaite pas privilégier à l'excès les échelons intercommunaux et régionaux. Très bien ! Nous y voyons un risque d'éloignement des organes de décision des territoires, à l'image de ce que nous avons défendu au sujet de la réforme des agences de l'eau. De cette même manière, certains points suscitent encore d'importantes interrogations, notamment en ce qui concerne l'Ademe. Nous ne comprenons pas, malgré les premières réponses apportées par la commission, sinon le sens, du moins l'intérêt de la réforme. En dernier lieu, je voudrais dire un mot de ce qui n'a pas été examiné dans ce texte. Un exemple nous a particulièrement affectés : durant ces deux semaines, nous avons souvent abordé la question des communes de montagne, ce qui n'a rien de surprenant dans un texte prônant la différenciation juridique des territoires. Mais, étonnamment, certains aspects n'ont pas pu être développés au motif d'irrecevabilités parfois peu compréhensibles. Notre collègue Guylène Pantel en a fait part durant les débats en indiquant regretter regretter que son amendement relatif au droit de l'urbanisme et aux risques d'une double application des lois Littoral et Montagne ne puisse être examiné. Dans ce même esprit, je pense à l'amendement qu'aurait souhaité porter notre collègue André Guiol visant à repenser les conséquences de la suppression des zones NB dans les règlements locaux d'urbanisme. L'ambitieuse simplification aurait justifié que ces sujets soient au moins abordés, tant ils sont l'objet, pour nos communes, de difficultés au quotidien. Aussi, au regard de ces éléments, vous comprendrez que le groupe du RDSE ne tiendra pas une position unanime.

Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, nous arrivons au terme de ces débats très riches, de ces dix jours et nuits passés ensemble, avec plus de 1 000 amendements examinés en séance. Je tiens à remercier la commission des lois, son président, François-Noël Buffet, et ses rapporteurs, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, qui ont accompli leur mission avec conviction.

Je souhaite aussi vous remercier, madame la présidente, ainsi que l'ensemble de vos collègues qui ont présidé pendant ces dix jours de séance, pour l'exigence d'efficacité et de sérénité que vous avez portée. Je veux souligner l'état d'esprit constructif dans lequel nous avons collectivement oeuvré et que nous partageons depuis de nombreux mois. Comme je le soulignais en ouverture de nos débats,

à ceux qui veulent réécrire l'histoire et faire passer le récit d'une confrontation- il n'en a rien été

Je retiens aussi qu'un grand nombre de mesures importantes ont été adoptées. Les différents orateurs qui se sont succédé les ont rappelées. Je ne vais pas être exhaustive, mais je voudrais retenir l'extension du pouvoir réglementaire local, la pérennisation de la loi SRU et sa mise en oeuvre différenciée le contrat de mixité sociale, le transfert des routes nationales aux départements et l'expérimentation en direction des régions volontaires, la capacité pour les collectivités à financer des établissements de santé et à recruter des soignants, l'expérimentation de la recentralisation du RSA ou encore le renforcement des pouvoirs des collectivités locales pour mettre en oeuvre concrètement la transition écologique sur leur territoire. Je ne serai pas plus longue : toutes ces mesures portent des avancées concrètes au bénéfice des territoires et de nos concitoyens. Je vous remercie de nouveau, toutes et tous, pour votre investissement et je remercie ceux d'entre vous qui ont voté en faveur de ce texte, qui répond aux besoins concrets des territoires. Mes chers

La séance est reprise.

L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020

Madame la présidente, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner, en nouvelle lecture, le projet de loi de règlement que vous

est exceptionnelle, en ce qu'elle témoigne de la réponse massive et rapide apportée par l'État à la crise que nous avons connue et qui s'est traduite par la mise en oeuvre d'un certain nombre de dispositifs nécessaires pour limiter l'impact économique des mesures prises pour protéger l'ensemble des Français. Ces mesures ont représenté un choc important pour notre économie et entraîné une récession de 7,9 %. Immédiatement après l'annonce du premier confinement, nous avons donné aux acteurs économiques les moyens de tenir bon. Avec le concours du Parlement, nous avons créé trois dispositifs de soutien dès le premier projet de loi de finances rectificative, renforcés et améliorés au fil du temps.

ont été versés en réponse à une dizaine de millions de demandes, portées par 2,2 millions d'entreprises. Je pense aussi aux prêts garantis par l'État. Ce dispositif a connu un succès important : plus de la moitié des entreprises des secteurs les plus touchés y ont eu recours et un tiers des entreprises a contracté un PGE, pour un total de plus de 140 milliards d'euros.

Au-delà de la question du financement, le résultat confirme que l'État a fait les bons choix : ces dispositifs ont permis de préserver le pouvoir d'achat des Français, qui a globalement augmenté de 0,4 % en 2020, malgré une baisse de production d'environ 8

Si l'exécution budgétaire a permis de soutenir l'économie en 2020, c'est aussi parce que nous avions reconstitué des marges de manoeuvre budgétaires depuis 2017. Je me dois de rappeler que le déficit public de 2019 a été le plus faible depuis 2001, retombant à 2,2 % du PIB, hors CICE.

pour les finances de l'État. Nous aurons l'occasion d'en débattre, et nos travaux seront nourris par d'autres initiatives, notamment celle de M. Jean-Marie Vanlerenberghe et de la commission des affaires sociales sur les lois organiques pour le financement de la sécurité sociale.

Ce projet de loi clôt budgétairement une année 2020 exceptionnelle à bien des égards, compte tenu bien évidemment de l'épidémie de covid-19 et de ses conséquences sur notre économie et sur l'économie mondiale.

Par ailleurs, cette année d'exécution exceptionnelle s'accompagne d'une dégradation d'une ampleur inédite de nos comptes publics, avec un déficit budgétaire de l'État d'un niveau tout aussi inédit de plus de 178 milliards d'euros. Chacun le sait, cette crise a rendu urgente et vitale la mise en oeuvre de mesures de soutien tant aux entreprises qu'aux ménages. Ainsi, plus de 40 milliards d'euros ont été dépensés sur la seule mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire », qui n'existait bien évidemment pas en loi de finances initiale. Le Sénat a voté ces mesures de soutien, qu'il s'agisse du fonds de solidarité, de l'activité partielle ou des PGE.

contraint à moins intervenir sur fonds publics, en recourant, par exemple, davantage aux prêts garantis par l'État qu'à des subventions directes. Il est regrettable de subir ainsi le choix du Gouvernement de reporter systématiquement le redressement des comptes publics au cours des dernières années, alors que l'on bénéficiait à la fois d'une croissance supérieure à son potentiel et d'un fort dynamisme des prélèvements obligatoires. Cette situation nous a indéniablement fragilisés lorsque la crise est survenue : nous payons maintenant les conséquences des choix pris par le Gouvernement, qui n'a pas su- ou voulu -créer les conditions qui nous auraient permis de disposer de marges de manoeuvre budgétaires supplémentaires, qui nous auraient été bien utiles.

Nous avons en particulier adopté les mesures de soutien qui étaient essentielles pour maintenir les entreprises à flot et protéger les ménages. Toutefois, nous ne partagions pas tous les choix du Gouvernement ayant guidé la construction de la loi de finances initiale pour 2020.

de première lecture. Par cohérence avec le vote du Sénat en première lecture, la commission propose à notre assemblée de ne pas adopter le projet de loi de règlement et d'approbation des comptes de l'année 2020

entièrement ces deux qualités. Je suis moi-même constant et persévérant dans mes efforts de pédagogie pour développer une gestion rigoureuse de l'argent public. Je pense que cette culture de la rigueur manque beaucoup dans notre pays et dans notre administration.

que nous avions portées avec les sénateurs et sénatrices du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans le cadre de notre contre-budget. Ainsi, nous avions proposé la création de nouvelles solidarités, avec la hausse du RSA, un plan pour l'hôpital et l'autonomie, l'augmentation de l'aide alimentaire, un plan en faveur des outre-mer, la prise en charge du chômage partiel à 100 %, un plan de soutien à la vie associative et un renforcement du plan de soutien au secteur culturel. Nous avions également proposé des moyens pour que notre jeunesse ne soit pas une génération sacrifiée au sortir de cette crise : création d'une dotation d'autonomie jeunesse ; prise en charge élargie des frais de scolarité ; financement de projets associatifs ou professionnels pour les jeunes. Nous souhaitions enfin que l'écologie et le développement durable soient davantage au coeur de la réponse à la crise, avec l'accélération de la conversion des transports polluants, le lancement d'un grand plan pour la ruralité, un financement supplémentaire pour l'isolation sonore des bâtiments

reports de l'année 2020 rendent très crédible le contre-budget que nous avions proposé à l'automne. Et je ne parle pas de ce qui aurait pu être fait pour mettre davantage à contribution ceux qui le peuvent, en particulier les bénéficiaires capital ! Pour notre part, nous considérons que l'approche du Gouvernement est insuffisante sur les questions environnementales et sociales, sur la solidarité et la préparation de l'avenir. Nous ne partageons pas cette idée

mais quand il y a une erreur de réglage, une erreur d'anticipation, cela conduit à des paris ratés.

aujourd'hui, nous jouons une partie dont nous connaissons déjà l'issue, puisque le Sénat a rejeté en première lecture le projet de loi de règlement

il est donc fort probable que la Haute Assemblée rejettera de nouveau le projet de loi de règlement pour 2020, les données du problème n'ayant pas changé. Le groupe Les Indépendants a déjà eu l'occasion de dire qu'une majorité de ses membres soutenait ce projet de loi, non parce qu'il comporte de bonnes nouvelles,

quelques points auxquels mon groupe, dans son ensemble, reste attaché. À l'heure où nous nous apprêtons à boucler les comptes d'un exercice budgétaire hors norme, il est important de fixer un cap clair pour nos finances publiques, car l'année 2020 l'année 2020 pèsera encore longtemps de son fardeau sur notre souveraineté économique. Nous comprenons la nécessité de relancer, au plus vite et au plus fort, l'économie, pour lui permettre de retrouver rapidement son rythme de croisière.

pour financer la sécurité sociale, l'Unédic, les retraites, il nous faudra renouer avec une forme de rigueur budgétaire. Le programme de stabilité semble, à cet égard, manquer d'ambition : la perspective d'un retour du déficit public sous la barre des 3 % n'est pas prévue avant 2027. Il s'agit non pas d'une obsession comptable, mais bien de notre capacité à fixer nos priorités politiques. Comment financer de nouveaux droits pour les jeunes, pour les jeunes, comme l'a annoncé le Président de la République, si nous ne sommes pas capables de contenir la hausse des dépenses dans d'autres domaines ? La rigueur budgétaire est d'abord affaire de priorités politiques. Pour nous, le sérieux budgétaire ne doit pas se faire aux dépens des missions régaliennes de l'État, comme l'éducation, la sécurité, le plan Santé, avec l'hôpital, et le plan Grand Âge. Âge. La crise économique ne devra pas non plus entamer notre action diplomatique, qui garantit l'influence française dans le monde, que ce soit par l'aide publique au développement ou nos capacités militaires. Au sein de nos frontières, nous devrons également veiller à préserver notre cohésion nationale, en repensant notre modèle social à partir de la valeur travail et de la valeur solidarité. Notre groupe soutiendra les mesures qui iront dans ce sens et votera en majorité pour ce texte. La

une inquiétude, largement partagée ici, sur la sincérité des choix budgétaires passés. Je ne reviens pas sur ceux, contestables, qui ont été faits par le Gouvernement pendant cette crise. Ils ont conduit à une réponse à la fois injuste et inefficace, ainsi qu'à la montée conjointe de la grande pauvreté et d'indécentes fortunes.

Je note également que les va-et-vient de flux financiers entre le budget de l'État et celui de la sécurité sociale ne laissent pas d'interroger. Il devient de plus en plus compliqué d'avoir une vision claire du financement de notre protection sociale, et je ne parle même pas de son autonomie ou de sa gestion avec les organisations du monde du travail. Je rappelle aussi les annonces, aides ou primes, qui ont été promises par le Gouvernement ou par le Président de la République, sans que l'on en voie encore la traduction budgétaire. Doit-on s'attendre pour le budget pour 2022 à une tonalité très électorale, voire électoraliste ? La seconde raison qui nous pousse à rejeter ce texte est une inquiétude plus vaste sur l'état des finances publiques. Il ne s'agit pas, comme sur certaines travées de cet hémicycle, d'être nostalgique du passé, de déplorer des taux d'endettement extraordinaires dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui des années 1970. Il ne s'agit pas non plus d'appeler à couper encore davantage dans nos services publics, ni à diminuer ce que vous appelez pudiquement les « dépenses de fonctionnement », et encore moins à affaiblir toujours davantage les outils et les moyens d'action de l'État. La problématique est tout autre elle se fonde non pas sur des lubies idéologiques, mais sur une réalité tragique. Le changement climatique, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans dix ans : c'était la semaine dernière, avec les canicules au Canada ou en Inde ; c'était ces derniers jours, avec les inondations en Allemagne, à Liège, en Chine ou dans le nord-est de la France. Notre responsabilité collective, c'est de tout faire, tout d'abord, pour atténuer ce changement climatique, car, s'il est bien trop tard pour l'empêcher, il s'agit d'en limiter l'ampleur et, ensuite, pour adapter nos sociétés à une augmentation inquiétante à plus de 2 degrés. Il y a là une autre forme d'insincérité que nous dénonçons. Nous savons parfaitement bien ce qui nous attend. Il vous suffit d'ouvrir les journaux de ce week-end, de lire les rapports qui vous sont destinés, à savoir ceux du GIEC et du Haut Conseil pour le climat. Il y a des faits : à ce jour, nous émettons 42 gigatonnes de CO2 par an. S'il est maintenu, ce chiffre nous fera dépasser inexorablement le seuil de 1,5 degré de réchauffement climatique dès 2031. Il nous faut donc impérativement réduire drastiquement ces émissions, et cela ne coûte pas si cher. D'après l'Institut de l'économie pour le climat, le coût serait de l'ordre de 1 % à 2,5 % du PIB par an. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Cela suppose de renforcer les moyens d'action de l'État, des collectivités, au lieu de les sous-estimer, voire de les délaisser, et de payer à prix d'or des expertises externalisées à des cabinets privés. Il est essentiel d'avoir des informations sur la qualité de la dépense publique au regard de cet objectif écologique. Pour cela, il est impératif de disposer d'une véritable comptabilité écologique et, bien sûr, de subordonner les aides publiques au respect de critères écologiques et sociaux stricts. Cessons ce gaspillage de dépenses inutiles

Je salue cet esprit de responsabilité, qui a permis d'apporter une réponse rapide et ferme à la crise. Seulement, le rejet de ce projet de loi de règlement du fait de l'abstention de la majorité sénatoriale et l'échec de la commission mixte paritaire viennent mettre fin à cette période d'union nationale.

Vous étiez à nos côtés, mes chers collègues, pour voter des crédits supplémentaires pour faire face à la crise tout au long de son évolution : 6,3 milliards d'euros dès le mois de mars 2020, pour répondre dans l'urgence à la première vague, puis 38 milliards d'euros au mois d'avril, 12 milliards d'euros en juillet et 19 milliards d'euros en septembre. Mais vous nous dites que le compte n'y est pas. C'est un peu facile Sur le fond, pourtant, nous partageons certaines de vos préoccupations, la situation d'ensemble des finances publiques étant inquiétante, et ce depuis des années. La crise est intervenue dans un contexte de solde dégradé de nos finances publiques et a conduit à une augmentation importante de la dette publique. En 2017, le Gouvernement avait entamé un chantier de redressement de nos finances publiques, le déficit passant même de 3,6 % en 2016 à 2,2 % en 2019, à la veille de la crise.

l'évolution de notre solde budgétaire est la conséquence de nos votes, qui ont permis d'apporter un soutien indispensable à nos concitoyens pendant la crise. Vient ensuite la question des crédits non consommés en 2020 et qui ont été reportés en 2021. La gestion de la crise sanitaire et la mise en place de dispositifs d'une ampleur inédite ont constitué un défi sans précédent pour le Gouvernement et pour nous, parlementaires, qui avons voté ces crédits. Les surbudgétisations, que certains d'entre vous ont pu souligner, ne sont pas le signe de l'insincérité de l'exécution budgétaire, elles témoignent plutôt de la prudence du Gouvernement et des prévisions sur lesquelles il s'est appuyé tout au long de la crise. Certes, ces sous-consommations sont importantes, mais n'oublions pas le contexte d'incertitude dans lequel nous avons voté ces enveloppes. J'ajoute que ces reports de crédits ne sont pas une surprise, puisqu'ils découlent de ce que nous avions décidé avec le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Mes chers collègues, alors que l'Assemblée nationale vient d'achever l'examen des propositions de loi organique visant à rénover le cadre de nos finances publiques, plus que jamais nécessaire de réformer la LOLF et de réfléchir à un meilleur pilotage financier de nos comptes publics, ainsi qu'à un renforcement du contrôle parlementaire en la matière. Nous ne pouvons juger l'année qui vient de s'écouler comme si rien ne s'était passé. Nous sortons de la crise la plus grave qu'a connue notre pays depuis la Seconde Guerre mondiale. À cette aune, nous pouvons reconnaître que la gestion budgétaire du Gouvernement a été sincère et prudente, compte tenu de toutes ces incertitudes. S'il faut aménager les règles organiques, c'est pour que la gestion rigoureuse de nos finances, lorsque la croissance est au rendez-vous, nous permette de soutenir le pays en temps de crise en répondant à la demande de nos concitoyens, de nos entreprises et des collectivités. C'est ce que nous avons fait et que nous continuerons à faire. Pour toutes ces raisons, et en cohérence avec l'ensemble des votes intervenus en 2020, le groupe RDPI votera une nouvelle fois ce projet de loi de règlement et invite tous ceux qui ont voté à nos côtés les quatre PLFR de crise à faire de même. La

On pourrait ajouter : sans savoir que la session parlementaire n'est pas encore achevée. Jeudi dernier, en première lecture, la majorité sénatoriale a laissé les oppositions de gauche rejeter le projet de loi de règlement du budget 2020. Je ne reviendrai pas en détail sur les raisons du rejet d'un texte essentiellement de constatation. Elles ont déjà été données. Cette nouvelle lecture offre au moins une occasion supplémentaire de débattre des questions budgétaires avant la suspension estivale, même si le temps imparti pour évoquer ce sujet assez technique est plus que limité. Depuis un an et demi, la crise du coronavirus a eu des conséquences énormes en matière sanitaire, mais aussi en matière sociale, économique et budgétaire. Alors que nous espérions pouvoir enfin tourner la page, la recrudescence des cas positifs laisse craindre le retour, plus rapide que prévu, de mesures de restriction, et ce malgré les progrès indéniables de la vaccination. Sur le fond, nous avons globalement approuvé les maintes révisions du budget l'an dernier. En cohérence, mon groupe a voté majoritairement en faveur de ce projet de loi de règlement, le montant important des reports de crédits en 2021. Cette législature devra assumer le surcroît inédit d'endettement public contracté en 2020-2021, dont l'impact devrait toutefois être nuancé, avec des taux d'intérêt historiquement bas et, peut-être, un léger retour de l'inflation. La hausse de l'endettement public depuis trente ans est, quant à elle, une responsabilité politique partagée par les différents camps. Il est vain de vouloir en attribuer à tel ou tel l'entière responsabilité. En revanche, c'est notre responsabilité et celle des gouvernements à venir d'y apporter des réponses convaincantes et acceptables par le plus grand nombre. Dans le budget exécuté en 2020, on constate à la fois le résultat des politiques menées les années précédentes et la rupture due à la crise sanitaire. On peut saluer un réel effort de « sincérisation » du budget et des hypothèses globalement raisonnables 2020 a été l'année où le déficit structurel s'est le plus approché de l'objectif de 0,5 % fixé par le traité européen sur la stabilité, la croissance et la gouvernance. En même temps, le déficit final s'élève à 178 milliards d'euros, quasiment le double de celui prévu par la loi de finances initiale, et il devrait être encore plus important en 2021. On discute beaucoup de montants et de quantités d'argent public, mais il faudrait aussi s'intéresser à la qualité de la dépense publique. En la matière, les indicateurs présentés dans le tome 2 du rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques, que je n'ai pas le temps de détailler ici, montrent que beaucoup de progrès peuvent encore être réalisés, qui concerne la qualité de la dépense pour l'usager que son efficience pour le contribuable. Pour anticiper un peu sur la rentrée, je précise que nous aurons bientôt l'occasion de débattre plus en profondeur de ces règles budgétaires,

contre le projet de loi de règlement.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera contre le projet de loi de règlement. C'est un exercice impropre. Je vais m'arrêter sur un phénomène d'ampleur : la privatisation de la gouvernance publique. Cet exercice budgétaire traditionnel vise à arrêter les normes financières et juridiques imposées à l'administration, donc les ressources dont dispose la puissance publique pour exercer ses missions.

le secteur public a perdu 180 000 agents entre 2006 et 2018. Il faut y ajouter 220 000 agents transférés des ministères vers les établissements publics,

Ce yo-yo politique a une histoire. Le non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux dans la fonction publique dans le cadre de la révision générale des politiques publiques en est une illustration. L'objectif est toujours le même : faire baisser l'emploi public pour tenter de faire baisser les dépenses, sauf que, sous couvert de maîtrise des dépenses publiques, on recourt à des acteurs parfois moins qualifiés et plus onéreux, ce qui aggrave la situation financière. Le recours à des cabinets privés en est réduit à payer deux fois des consultants : la première pour l'aider à faire des économies ; la seconde pour suppléer aux carences que ces mêmes consultants ont contribué à organiser. Tout y passe : organisation, management, santé publique. En tout, ce sont 500 contrats passés en trois ans. veille de l'examen d'un texte sur ce sujet fondamental, le pilotage de la crise sanitaire n'échappe pas à ce phénomène profond. Sur les dix premiers mois de la pandémie, vingt-six contrats ont été conclus avec ces cabinets. Qui prend les décisions ? En tout état de cause, les responsabilités du Président de la République et de son gouvernement sont engagées. On nous parle dorénavant d'adapter « des », et non pas « nos », outils de gestion de crise sanitaire, déjà choisis et peu débattus. Le texte modifie ceux sur la sortie de la crise et la prorogation de l'état d'urgence. Crise et état urgence deviennent donc des outils, dénommés adaptations. En bref, il s'agit d'organiser la division par la normalisation d'une situation exceptionnelle. La crise appelle des solutions et pas seulement des adaptations. C'est cruellement vrai avec la santé, secteur qui a le plus pâti d'une privatisation désarmante face au covid. des acteurs majeurs de la gestion de la pandémie. Nous en avons souvent débattu dans l'hémicycle. Chargées de coordonner la politique de santé au niveau local, elles constituent un moyen d'imposer austérité et contraintes au secteur hospitalier. En 2017, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes s'interroge sur la façon de mutualiser les établissements privés et publics. En 2018, elle débourse 300 000 euros pour du coaching. En 2020, quatre ARS commandent au privé une analyse de la situation financière des établissements de santé de leur région. Et la liste est longue, comme l'ont si bien détaillé le collectif « Nos Services Publics » et un très bon dossier dans ! La privatisation de leurs missions contribue à affaiblir la puissance publique, qui perd en compétences, en savoir-faire et en expertise. Le cercle est vicieux,

lois de règlement. Comment justifier cette abstention ? D'une part, nous relevons que, dans la durée, le Gouvernement a renoncé à redresser significativement

être conjoncturelles se trouvent désormais prises en compte dans le déficit structurel. D'autre part, ainsi que le rapporteur général l'a bien dit, l'extrême prudence du Gouvernement s'est transformée en une sorte de mépris du Parlement.

sont donc les raisons pour lesquelles le groupe Les Républicains s'abstiendra une nouvelle fois ce soir, entraînant très certainement le rejet du texte. La

7. Je vais mettre aux voix l'article 8. Je rappelle que, si cet article n'était pas adopté, il n'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble du projet de loi, dans la mesure où tous les articles qui le composent auraient été rejetés.

je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire, puisqu'il n'y a plus de texte. En conséquence, le projet de loi de règlement